La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, modifié par lettre rectificative, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

de nombreuses collectivités sont propriétaires de ces sites -ou privés des conventions de gestion, au travers desquelles elle se substituait à eux du point de vue de la responsabilité. Cependant, la Fédération, se trouvant dans l'impossibilité d'assurer financièrement l'augmentation importante de la prime d'assurance exigée, a dénoncé l'ensemble de ces conventions de gestion. des derniers mois, de nombreux sites ont donc été fermés, du fait des risques de recours. Les collectivités, qui sont très majoritairement propriétaires de ces sites, sont dans l'attente d'une simplification et d'une législation plus sécurisante

de cet amendement, il est proposé de limiter expressément la responsabilité du gardien d'un espace naturel au travers de l'acceptation par le pratiquant d'un risque inhérent à l'activité sportive concernée. Ce dispositif permet d'alléger la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires des sites naturels, tout en responsabilisant les usagers. L'objet de cet amendement a été particulièrement bien expliqué par notre collègue Savin. Il porte sur la responsabilité civile applicable aux propriétaires de sites naturels ouverts au public. Vous avez raison, mon cher collègue, il faut aujourd'hui légiférer.

Monsieur Savin, votre amendement porte sur la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires des sites naturels ouverts au public. Au travers de cette disposition, la responsabilité du gestionnaire de site naturel ne pourrait pas être engagée en cas de dommages causés aux pratiquants, si « ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque inhérent à la pratique sportive considérée ». Bien que le Gouvernement soit favorable à l'atténuation du régime actuel de responsabilité, afin de favoriser le développement de la pratique, il ne saurait soutenir une exonération aussi large, dans le cadre de la pratique d'un sport de nature. Il aurait été préférable que la responsabilité soit limitée aux risques « normalement prévisibles ». L'appréciation de la normalité et de la prévisibilité du risque permet en effet de tenir compte du comportement de ceux

s'appliquerait à toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé au sein desquelles, en vertu de la loi, des élus locaux agissent en qualité de mandataires de leur collectivité territoriale ou de leur groupement de collectivités territoriales. ne vise pas la situation des entités dénuées de personnalité morale, comme les régies dotées de la seule autonomie financière, dès lors qu'un conflit d'intérêts ne saurait naître en l'absence de personne morale extérieure à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales.

les associations ou groupements d'intérêt public que sont les missions locales ou les maisons de l'emploi, les établissements publics locaux à caractère industriel et commercial que sont les offices publics de l'habitat et, plus généralement, toutes les structures de droit public ou de droit privé pour lesquelles la loi prévoit la participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Dans ce cas de figure, la présente

ni au sens du code pénal qui prévoit une possibilité de délit de prise illégale d'intérêts. Les dispositions de cet amendement précisent toutefois les cas de figure dans lesquels les élus locaux seront amenés à se déporter, afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêts ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégation de service public, lorsque la personne morale est candidate, ni aux délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne morale ou portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette L'amendement vise également à prévoir une clause de réciprocité permettant, par symétrie, aux élus locaux agissant comme mandataires de leur collectivité territoriale ou de leur groupement dans des organismes extérieurs de ne pas être non plus considérés comme intéressés à l'affaire, lorsqu'ils sont amenés à délibérer dans le cadre de ces organismes au sujet de leur collectivité ou de leur groupement.

Cet amendement vise à clarifier, en les renforçant, les dispositions actuelles du CGCT, qui permettent à un élu local représentant la collectivité ou le groupement actionnaire au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise publique locale (EPL) de participer aux délibérations de l'assemblée délibérante, lorsque celle-ci statue statue sur ses relations avec cette EPL. Ces élus ne peuvent d'ores et déjà pas participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégation de service public de la collectivité territoriale ou du groupement, lorsque la SEML est candidate. Il y a lieu de préciser qu'ils ne peuvent pas non plus participer aux délibérations accordant une aide économique à la SEML, pas plus qu'aux délibérations les désignant ou leur assurant une rémunération. Par ailleurs, les élus locaux siégeant au conseil d'administration ou de surveillance de la société ne sauraient être exposés au même risque de conflit d'intérêts, par souci de réciprocité.

: la responsabilité des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour siéger soit dans une EPL, soit dans d'autres organismes, comme les missions locales ou les maisons de l'emploi.

large, parce qu'un élu désigné par sa collectivité pour la représenter au sein d'un organisme peut être accusé de prise illégale d'intérêts, dès lors qu'une décision prise par cet organisme

L'objet du présent amendement est de modifier la définition du conflit d'intérêts fixée à l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013, afin d'exclure de cette définition l'interférence entre deux intérêts publics, lorsque l'agent public ou l'élu concerné agit ès qualités dans le cadre d'une habilitation législative et dans l'exercice d'une activité pour laquelle il a été régulièrement élu ou désigné. Dès lors

l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Ce texte définit le conflit d'intérêts comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui surveille ces questions avec une attention toute particulière, signalait, dans son rapport d'activité de 2017, que le « conflit d'intérêts entre deux intérêts publics [ ...] constitue une exception au regard de l'appréhension internationale de cette notion. » La Haute Autorité avait donc proposé de « supprimer la possibilité d'un conflit entre deux intérêts publics ». Le présent amendement vise donc à préciser qu'il n'y a pas de situation de conflit d'intérêts entre deux intérêts publics, lorsque le membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale a été désigné pour siéger

à M. Christian Klinger. Cet amendement vise à mieux encadrer juridiquement la notion d'interférence entre les fonctions publiques et les intérêts privés du décideur public.

à la notion d'« intérêt quelconque » celle d'« intérêt personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public

à l'un des candidats avec une intention délibérée- cela revient à réintroduire l'élément intentionnel -et que cet avantage a directement conduit à lui attribuer le contrat de la commande publique. Quel

des prestations au profit de personnes non actionnaires de la société, en accord avec la réglementation européenne. Toutefois, les modalités de calcul du seuil de 80 % sont incertaines, notamment en ce qu'elles peuvent viser le chiffre d'affaires ou les coûts supportés, et pourraient donc donner lieu à interprétation devant le juge. La rédaction proposée, en faisant notamment référence à une « estimation réaliste », ne permet pas d'éviter cet écueil. Pour des raisons de sécurité juridique, notamment pour les élus concernés, il est nécessaire de maintenir la règle selon laquelle l'activité des SPL doit être réalisée dans son intégralité au profit des collectivités et groupements actionnaires. C'est pourquoi nous prévoyons prévoyons la suppression de l'article 73 Quel

exprimé par les EPL et de nombreuses collectivités. Toutefois, mon cher collègue, la disposition est très encadrée, puisque nous avons repris la définition stricte de la quasi-régie entre les collectivités

Je rappelle que les SPL ne concernent que des collectivités territoriales ou des personnes publiques et qu'il me semble hasardeux,

pour explication de vote. Je suis très défavorable à cet amendement. Contrairement à ce qu'a dit Mme la ministre, cette flexibilité est parfois utile dans le cadre des SPL. Je rejoins la position de Mme la rapporteure : de temps à autre,

la commission des lois propose de confier de nouvelles missions d'évaluation des politiques publiques territoriales aux chambres régionales des comptes. Le rapport de la commission fait référence à la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des communes, départements et régions, qui a institué les chambres régionales des comptes, bien connues des élus,

de la Cour des comptes dont elles assurent le maillage territorial -ont principalement trois compétences pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics : le jugement des comptes et comptables publics, le contrôle des comptes et de la gestion, le contrôle des actes budgétaires sur

commission est particulièrement utile pour faire évoluer les missions des chambres régionales des comptes et donner la faculté aux régions et départements de demander aux chambres régionales des comptes de leur ressort de procéder à l'évaluation d'une politique publique. Ce sera un appui important pour mener à bien des politiques publiques de plus en plus nombreuses et complexes, comme l'a rappelé

une difficulté quant à leur participation. Lorsque l'un d'entre eux est absent, il n'est pas possible d'organiser son remplacement par un autre parlementaire du département. Aussi, le présent amendement a pour objet, non pas de renforcer le pouvoir des parlementaires dans cette commission, mais de modestement le maintenir en cas d'absence à l'une des réunions. Il vise à permettre au parlementaire absent de désigner un autre député ou sénateur du département afin qu'il le supplée pour la durée de la réunion.

C'est le président du Sénat qui désigne les représentants du Sénat pour les départements comportant cinq parlementaires ou plus. Ceux-ci sont donc nommés par leurs assemblées pour siéger à la commission.

surcharger les collectivités d'obligations et d'investissements complémentaires. Si la commission comprend bien l'intention des auteurs de cet amendement, il lui semble que beaucoup de collectivités

Merci,

n'ayez pas transposé ou défiguré mes propos, je pense que nous sommes tous d'accord avec la nécessité de renforcer la transparence et l'information.

de 20 000 habitants et plus, comme cela est possible pour les régions, les départements et les communes de plus de 50 000 habitants. Le principe proposé me semble une excellente idée,

aujourd'hui rendu applicable aux EPCI à fiscalité propre par renvoi de l'article L. 5211-1. Or ce dernier article précise que ses dispositions sont applicables aux EPCI de plus de 50 000 habitants. La rédaction ne va donc

La loi prévoit une possibilité de révision libre qui implique les délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes

Le présent amendement a pour objet de préciser cette règle de majorité nécessaire à l'application de la procédure de révision libre des attributions de compensation lorsque cette procédure est engagée par délibérations concordantes de l'EPCI et des communes concernées. Il vise à préciser que la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil communautaire devant adopter la révision libre de l'attribution de compensation s'entend de la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Quel est l'avis de la commission

parole est à Mme la ministre. Le code général des collectivités territoriales prévoit aujourd'hui que les ministères porteurs d'un projet de texte réglementaire doivent transmettre des éléments d'information complémentaires ou une version modifiée du projet

En effet, si le CNEN est systématiquement saisi des projets de loi concernant les collectivités territoriales, contrairement à l'ancienne Commission consultative d'évaluation des normes d'un second examen après un premier avis défavorable du CNEN, dont la constitutionnalité n'est pas garantie, ralentirait le processus normatif. Cette modification n'est d'ailleurs pas demandée par les membres du CNEN. Il revient au Parlement, le cas échéant, en s'appuyant sur l'avis du CNEN, de modifier par amendement le projet de loi dans le cadre de la discussion parlementaire. Ce relais peut d'ailleurs être opportunément assuré par les représentants du Sénat siégeant au sein du CNEN.

ou d'une commission permanente d'une des deux assemblées peut demander au CNEN de formuler un avis sur un projet de loi afin d'en apprécier la pertinence au regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Il me semble que cet article confond le rôle du Conseil national d'évaluation des normes et

de vote. Madame la rapporteure, le choix de la libre administration des collectivités territoriales est déjà un choix politique.

est incidemment dépendante pour le rendu de ses avis des remontées de terrain des élus locaux émanant des différents échelons territoriaux, et ce afin d'éclairer les ministères porteurs sur les éventuelles difficultés d'application des projets de texte présentés.

divisé par deux en cours de mandat, au gré des élections locales et des démissions, sans possibilité de remédier à cette situation qui fragilise la légitimité

de faire évoluer dans le sens d'une plus grande souplesse, et dans un souci de simplification, la partie législative du CGCT afin de garantir non seulement la continuité, mais surtout la représentativité de l'instance, pendant l'entièreté du mandat de trois ans de ses membres. Le présent amendement vise donc à poser le cadre juridique du remplacement, en cours de mandat, des membres du CNEN, y compris des membres représentant l'État.

pour le rendu de ses avis des remontées de terrain des élus locaux émanant des différents échelons territoriaux, et ce afin d'éclairer les ministères porteurs sur les éventuelles difficultés d'application des projets de texte présentés. Or, en l'état du droit, cette représentativité n'est pas garantie durant l'entièreté du mandat qui est de trois ans, avec le risque de mettre en péril la légitimité des avis rendus par le CNEN. Il apparaît opportun de faire évoluer, dans le sens d'une plus grande souplesse, et dans un souci de simplification, la partie législative du CGCT afin de garantir non seulement la continuité, mais surtout la représentativité de l'instance, pendant l'entièreté du mandat de trois ans de ses membres. Le présent amendement vise donc à poser le cadre juridique du remplacement, en cours de mandat, des membres du CNEN, y compris des représentants de l'État. représentants de l'État. Il s'inscrit dans la droite ligne de la philosophie du Sénat visant à laisser davantage de marges de manoeuvre aux associations nationales d'élus dans la nomination de leurs représentants au sein des instances consultatives, comme en témoignent les amendements adoptés dans le cadre de la loi Engagement et proximité. Cette rédaction, mettant au coeur du processus de nomination les associations nationales d'élus, s'inspire des dispositions législatives en vigueur concernant le Comité des finances locales. Quel est l'avis de la commission

touristique, à l'agriculture, à l'environnement ainsi qu'à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.

autorisé sur la nécessité d'adapter toute nouvelle norme envisagée par les pouvoirs publics, conformément à l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 : « Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l'urbanisme, à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l'agriculture, à l'environnement ainsi qu'à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.

paraît justifier que les avis du CNEN, en l'espèce sur les propositions de loi, ne soient pas rendus publics. Et nous ne voyons pas pourquoi il faudrait appliquer un régime de publicité différent selon que l'auteur du texte est le Gouvernement ou un parlementaire.

Pour éviter un tel contournement, rendons publics les avis du Conseil national d'évaluation des normes, qu'il s'agisse d'un projet de loi ou d'une proposition de loi

publics de coopération intercommunale.

: La parole est à M. Jérôme Durain. Cet amendement tend à supprimer la mention qui permet à un parlementaire de s'opposer à ce que sa proposition de loi soit transmise pour avis au Conseil national d'évaluation des normes. Le Sénat, vous le savez, examine de nombreuses propositions de loi concernant les collectivités territoriales. parfois à vide, malheureusement, dans la mesure où, s'agissant de propositions de loi, nous ne disposons ni d'étude d'impact, ni d'avis du Conseil d'État, ni d'avis du Conseil national d'évaluation des normes. De tels avis d'organismes extérieurs seraient de nature à éclairer et à approfondir nos échanges, les rendant plus fructueux.

Actuellement, le Conseil national d'évaluation des normes n'est obligatoirement consulté que sur les projets de loi. Cet amendement vise à ce qu'il soit également obligatoirement saisi des propositions de loi, dès lors que celles-ci sont inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée. Ainsi n'aurait-il pas à examiner toutes les propositions de loi, mais uniquement celles dont nous serions amenés à discuter. Dans cette hypothèse, le CNEN disposerait d'un délai de deux semaines

: La parole est à M. Max Brisson. Cet amendement de Cyril Pellevat tend à permettre la saisine du Conseil national d'évaluation des normes par le président de la commission permanente d'un comité de massif

des caractéristiques différentes. Il s'agit de surcroît d'étendre le périmètre des demandes d'avis aux dispositions législatives, et non plus seulement réglementaires, mais uniquement lorsque la demande émane du Gouvernement, des présidents des commissions permanentes du Parlement ou du président du CNM.

Mercier, pour présenter l'amendement n° 213 rectifié . Les impôts directs locaux relèvent désormais exclusivement des communes et intercommunalités à fiscalité propre. Il apparaît plus que nécessaire et légitime d'associer leurs représentants aux travaux des commissions départementales des impôts directs.

J'ai eu l'occasion de présenter beaucoup de textes relatifs au droit funéraire. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'il s'agit, dans ces circonstances où les familles sont éprouvées, donc vulnérables, de les défendre,

d'une information actualisée, donc claire, transparente et fiable, il faut que nous prévoyions cette actualisation annuelle des sommes indiquées sur ces devis types. Voilà pourquoi il vous est proposé de compléter la loi de 2008 par cet ajout

je souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur cette proposition qui me semble aller dans le bon sens- mais j'aimerais m'assurer que la commission pense juste. Quel est Cet amendement a pour objet d'imposer l'actualisation annuelle des devis modèles obligatoirement déposés par les opérateurs funéraires dans certaines communes aux fins de libre consultation les familles des défunts. La consultation des devis modèles en mairie doit garantir au « consommateur » toute la clarté nécessaire concernant les prestations proposées par les opérateurs funéraires. Conscient que le dispositif actuel de mise à disposition des devis modèles par les communes présente de réelles difficultés de mise en oeuvre, le Gouvernement travaille actuellement à le moderniser.

choix éclairé. Je comprends aussi que votre souhait est de rendre le dispositif actuel plus contraignant sans pour autant traiter la question de son efficacité, qui est selon moi à la source des difficultés d'application rencontrées aujourd'hui.

du Gouvernement en la matière. Le projet de loi présenté par le Gouvernement prévoyait, dans son article 56, que l'ensemble des délégations octroyées aux conseils de territoire de la métropole feraient l'objet d'un réexamen par le conseil métropolitain trois ans après son renouvellement. Aux termes de cet article, le conseil métropolitain pouvait décider à cette occasion de mettre fin à ces délégations. L'objectif du Gouvernement, vous l'avez compris, était de permettre à la métropole de rééquilibrer la répartition des compétences en sa faveur au sein du niveau métropolitain, qui comporte un échelon territorialisé, les conseils de territoire. Il s'agissait de renforcer sa capacité à agir concernant des compétences stratégiques qui doivent être exercées à son niveau. Après échanges avec les acteurs locaux, le Gouvernement a décidé de soumettre au débat un amendement plus complet, tendant à dessiner un chemin faire sortir des blocages institutionnels. En effet, je me suis rendue à Marseille en mai dernier ; j'y ai rencontré de nombreux acteurs locaux des Bouches-du-Rhône, la présidente de la métropole, bien sûr, le maire de Marseille,

-a permis de dépasser les frontières administratives et de créer un cadre d'action pour traiter à la bonne échelle des sujets essentiels pour les habitants comme ceux des mobilités, du logement et de l'habitat, du développement économique et de l'attractivité. Malheureusement- tous les acteurs locaux le reconnaissent -, cette métropole est entravée dans son efficacité, car les compétences n'y sont pas toujours positionnées au bon niveau. Quant à ses moyens financiers, ils sont contraints par des décisions prises dans le passé, qui l'ont bridée. Il est temps de sortir de cette situation de blocage. Il existe aujourd'hui un consensus pour mettre fin au, bien que la méthode souhaitée par les différents acteurs ne soit pas toujours la même, je le reconnais, mais un dialogue s'est ouvert et il nous est possible de faire bouger les lignes, car les intéressés y sont prêts. Je remercie les sénateurs des Bouches-du-Rhône, qui y travaillent.

En premier lieu, il est nécessaire de faire redescendre des compétences de proximité au niveau des communes lorsque leur exercice à cet échelon peut contribuer à une plus grande efficacité de l'action publique. Un consensus important s'est exprimé sur ce sujet depuis le rapport du préfet Dartout. Je propose ainsi que la métropole puisse restituer aux communes qui le souhaitent des compétences relatives aux parcs et aires de stationnement, aux crématoriums, ainsi qu'au service public de défense extérieure contre l'incendie.

serait satisfaite une attente de l'ensemble des acteurs locaux sans remettre en cause les mutualisations existantes. En deuxième lieu, nous devons redéfinir la répartition des compétences entre la métropole et les conseils et les conseils de territoire. La métropole doit pouvoir exercer les compétences stratégiques d'une grande métropole en matière de transport, d'aménagement, d'habitat et de développement économique. En troisième lieu, afin de préserver l'ancrage territorial de la métropole, les prérogatives spécifiques de la conférence métropolitaine des maires seront élargies. Enfin, nous devons aller vers un nouveau calcul des attributions de compensation, qui soit plus juste et plus approprié aux compétences effectivement transférées, et qui redonne à la métropole des moyens d'action.

c'est-à-dire à la recherche d'une coconstruction avec les élus locaux ; je souhaite poursuivre ce travail avec vous. Je partage votre volonté de trouver des solutions pour faire bouger la répartition des compétences Vous savez que je ne partage pas la méthode que vous proposez, mais il est toujours possible d'avancer et de discuter. En effet, il ne me paraît pas souhaitable de figer dans le temps les délégations de compétences aux communes sans décider quelles sont celles qui devraient être définitivement restituées.

qui est, comme on le dit souvent, la porte de la France sur la Méditerranée. C'est donc dans un esprit absolument constructif que le Gouvernement a déposé l'amendement

difficile pour de nombreux maires de maîtriser le destin de leur commune. C'est d'autant plus vrai que la métropole n'a pas vocation à exercer les à exercer les compétences de proximité- elle n'en a pas les moyens. Je salue d'ailleurs la volonté du Gouvernement

Je rappelle en effet que, pour engager une telle réforme, nous devons revenir à l'esprit originel de l'intercommunalité et laisser les élus définir le plus librement possible les compétences stratégiques ou opérationnelles qu'ils souhaitent partager. Les communes membres de cette métropole doivent avoir la liberté de s'organiser en fonction

à la carte entre les communes et la métropole. En tout état de cause, madame la ministre, faisons confiance à l'intelligence collective locale pour décider d'une nouvelle répartition plus efficace des compétences, en confortant la métropole dans l'exercice de ses compétences stratégiques et en

le problème connu, repéré, identifié, étudié, notamment par le préfet Dartout, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence : inefficace, inopérante, peu attractive- je partage le constat et de Mme Gourault et de M. Le Rudulier. Cette métropole est née dans la douleur ; son acceptabilité par les communes a toujours fait défaut, il faut le savoir ! Elle portait en elle dès sa création plusieurs problèmes qui n'ont, à la surprise de personne, pas plus trouvé de solution pendant l'ère de M. Gaudin qu'après le changement politique survenu à la tête de sa ville-centre, Marseille, voilà quelques mois. La gouvernance pose problème. Par exemple, comment justifier que la personne qui dirige la métropole cumule la responsabilité de l'exécutif départemental avec celle de son équivalent métropolitain, alors même qu'elle n'a pas su convaincre les électeurs de la ville-centre de Marseille

pour mettre en commun le destin d'un territoire en confiant à l'échelon métropolitain des compétences structurantes et stratégiques, que nous approuvons, n'est en rien en opposition avec l'exercice de compétences de proximité par l'échelon qu'est la commune Au sein de la métropole, cette volonté de conserver ces compétences de proximité a été autorisée des délégations ou par un délai accordé pour transférer ces compétences à la métropole pour certaines communes.

Je vous remercie

par M. Le Rudulier visant à donner à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à ses communes membres les moyens de clarifier la répartition de leurs compétences. En fin de semaine dernière, le Gouvernement a déposé très tardivement un amendement visant à réécrire intégralement cet article 56. Très dense, l'amendement du Gouvernement peut s'analyser en trois parties. La première partie correspond à une demande que nous faisions depuis longtemps, à savoir la restitution aux communes de certaines compétences de proximité. La deuxième partie allonge la liste des compétences métropolitaines non délégables aux conseils de territoire. Enfin, la troisième partie aménage une procédure dérogatoire visant à contraindre les communes de la métropole à une baisse de leur attribution de compensation, à la majorité simple et en faisant éventuellement appel à la chambre régionale des comptes, qui sortirait, de fait, totalement du rôle régalien qui est le sien pour l'ensemble des collectivités françaises. Concernant la métropole d'Aix-Marseille-Provence, il n'est pas anodin de savoir qu'un territoire possède à lui seul 54 % des voix et que les cinq autres conseils de territoire pourraient se voir contraints, sans qu'une réelle consultation ait lieu, à des baisses mettant leur budget en réelle difficulté. Certaines communes ne seraient plus à l'équilibre. Cette simple constatation montre que la précipitation, madame la ministre, dans le désir d'une réforme n'est jamais la bonne solution. Le Gouvernement a montré par cet amendement que la métropole d'Aix-Marseille-Provence méritait une attention particulière en raison de son étendue, de ses spécificités et de la diversité des territoires qui la composaient. Certes, c'est une avancée importante et une ouverture vers les négociations à venir, qui doivent se faire avec les élus locaux, lesquels ont entamé une réflexion en profondeur sur la se faire avec les élus locaux, lesquels ont entamé une réflexion en profondeur sur la réforme nécessaire de l'institution métropolitaine. Enfin, il est important que le Gouvernement se rapproche des maires. Proposer une réforme de cet EPCI

conclues entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et ses conseils de territoire pour l'exercice de certaines de ses compétences afin de répondre à l'insatisfaction des élus locaux sur l'organisation actuelle. Les modifications apportées par la commission des lois n'étaient pas de nature à satisfaire les tractations en cours entre le Gouvernement et la métropole, notamment sur le montant des attributions de compensation versées par la métropole à ses communes membres. L'amendement n° 1734 rectifié du Gouvernement vise à pallier cette difficulté en limitant les possibilités de délégation des compétences aux conseils de territoire, en complétant la liste de celles qui ne sont pas délégables et en ouvrant la possibilité de restituer plusieurs compétences de proximité aux communes membres lorsque leur exercice à cet échelon contribue à une plus grande efficacité de l'action publique. Bien que cette proposition ne semble pas fédérer l'ensemble des travées du Sénat, le groupe RDPI votera en faveur de cet amendement pour trois raisons : la réponse aux attentes des élus locaux de la métropole la recherche de compromis engagée par le Premier ministre et par Mme la ministre ; et surtout la souplesse accordée par le Gouvernement en matière de compétences, ce qui n'a jamais été proposé auparavant. La parole est à M. Jérémy Bacchi,

À ce titre, les premières années de fonctionnement de la métropole nous amènent à souhaiter quelques ajustements : c'est le cas, notamment, des compétences « de proximité », dont l'exercice s'avérerait plus efficace pour certaines d'entre elles si elles étaient redéléguées aux communes. De premiers échanges entre les parlementaires du département, les élus communaux et intercommunaux, mais aussi avec l'association des maires du département, ont permis d'affiner des propositions pour une meilleure articulation commune-métropole. Il est en effet indispensable de sortir du fonctionnement actuel particulièrement illisible, juridiquement instable et lourd administrativement, car sous-tendu par 208 conventions de gestion. Pendant des décennies, notre territoire s'est construit sur une opposition parfois savamment entretenue entre Marseille, d'un côté, et le reste du département, de l'autre. Il est grand temps de dépasser ces querelles stériles et d'oeuvrer ensemble au développement de notre territoire tout entier. Même si les communes doivent être l'échelon de proximité, nous le disons avec force, il est important de souligner le rôle essentiel joué par les conseils de territoire. Cet échelon intermédiaire entre la métropole et les communes constitue un rouage de l'action territoriale particulièrement adapté pour traiter les problématiques spécifiques à chacun des bassins de vie et d'emploi très divers qui constituent ce vaste ensemble qu'est la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Au sein de ces conseils de territoires, il est néanmoins fondamental que chacune des communes-centres soit pleinement représentée et dispose de prérogatives pour orienter au mieux l'action publique et répondre aux besoins de ses administrés. Cela doit être notamment le cas pour la commune de Marseille, deuxième ville de France, dont la représentation au sein des instances du conseil de territoire Marseille-Provence doit être reconsidérée et repondérée. Oui, nous avons besoin d'une métropole, mais d'une métropole de projet, d'une métropole qui se recentre sur ses compétences essentielles telles que les transports, le développement économique, les questions environnementales. Pour le reste, les communes doivent retrouver leurs compétences, cela a été dit avant moi sur les travées de cette assemblée, assemblée, de proximité ou,, les déléguer aux conseils de territoire, échelons intermédiaires et plus efficients. Je pense notamment aux compétences de voirie

dès son accouchement, car c'est une des métropoles qui a mis le plus de temps à voir le jour. C'est aussi une des métropoles qui a, peut-être avec le temps, éloigné le plus le processus de décision,

à l'urgence de la situation. On ne peut plus fonctionner avec 208 conventions de gestion : c'est impossible ! Ensuite, c'est aussi un amendement qui remet l'élu, singulièrement les élus municipaux, au coeur du processus de décision

Nous l'avons suffisamment dit et reproché, il existe un véritable problème avec les études d'impact accompagnant les projets de loi présentés par le Gouvernement. Comment voulez-vous

Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises en commission des lois, beaucoup de métropoles, parce qu'il est finalement devenu « cosmétique » de demander sa métropole, n'exercent pas leurs pleines compétences. Il faudra assez vite revenir devant le Parlement pour traiter de cette problématique métropolitaine.

: La parole est à M. Guy Benarroche. Pourquoi s'opposer à cet article tel qu'il a été réécrit par le Sénat ? Cette réécriture sécurise légalement les délégations de compétences qui ont été condamnées récemment à la suite d'un recours gracieux du préfet. Elle maintient également et étend la possibilité pour les communes ayant conservé leurs compétences de ne pas les faire remonter à l'intercommunalité, c'est-à-dire à la métropole ou à ses conseils de territoires. Pourquoi alors s'y opposer ?

1 (CT1). Ces communes-là qui avaient transféré leurs compétences de proximité, comme la voirie de proximité, en particulier à Marseille, ne pourront pas les récupérer alors qu'elles le demandent depuis des mois et des années. Loin de vouloir faire de Marseille une ville spéciale par sa taille ou son rôle de ville-centre- je vous rappelle qu'elle représente 48 % de la population de la métropole d'Aix-Marseille-Provence

les problèmes de gouvernance, les problèmes de mode de scrutin, les problèmes de périmètre de la métropole et des conseils de territoire, les problèmes de ressources financières ne sont pas traités

Chacun reconnaît, un peu comme pour le Grand Paris, que cette situation ne peut pas rester en l'état, d'autant qu'il existe un problème juridique

une infrastructure miraculeuse, dont tout le monde serait content, qui fonctionnerait bien et qui serait pérenne, relève non pas d'une ambition, mais d'une folie hors de portée ! Quand le précédent gouvernement s'est exercé à créer la métropole de Marseille, on a vu le genre d'inventions qu'on a eu

permettre une territorialisation de compétences à la carte, j'y reviendrai, car c'est absolument génial, c'est ce que le Sénat demande depuis cinq ans et que vous lui refusez ... Deuxièmement, sur l'attribution de compensation, vous affirmez qu'il y aura deux possibilités pour la métropole de Marseille de revoir l'attribution de compensation. La métropole pourra notamment saisir la chambre régionale des comptes, qui étaye son appréciation sur les attributions de compensation versées aux communes et fixera un nouveau montant qui s'imposera,

qui est une métropole générique, à laquelle s'appliquent quelques dispositions particulières, vous ouvrez le droit, car il y a nécessité et besoin, à la définition de l'intérêt communautaire et à la territorialisation.

institutionnel de répartition des compétences. J'ajoute un point qui me paraît essentiel pour tendre de nouveau la main au Gouvernement : dès le mois de juillet 2020,

que les cinq autres EPCI ont conservé la voirie à l'échelon communal. On voit bien que cette métropole à la carte est nécessaire sur certaines

un destin commun, sans même prendre le temps de le construire. Finalement, une des réponses- et c'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas la suppression de cet article -, c'est d'acter cette réalité, tout en renforçant

pour la métropole de Marseille. Vous le savez bien, en l'état actuel des choses, que nous votions l'amendement du Gouvernement ou que nous adoptions l'article tel que vous l'avez bâti, monsieur Le Rudulier,

Il faut rendre les compétences de proximité aux maires, c'est-à-dire à ceux qui savent et savent faire. Ces maires qui, pour la très grande majorité d'entre eux- pour ne pas dire tous ou presque tous -, sont au fait de ce dont leur commune et leurs administrés ont besoin. Je pense en particulier aux logements sociaux, synonymes de contraintes idéologiques ou de sanctions financières. Je rappellerai aussi cette phrase d'un cynisme absolu prononcée par Christian Eckert, alors ministre du budget du président Hollande : « La fusion des régions a été décidée pour contrer le Front national. Autant dire qu'elle a été décidée contre l'idée démocratique et l'efficacité de gestion ... Au moins, cela avait le mérite d'être assumé ! Le système politique, tous bords confondus, se replie dans ses citadelles de mépris et réforme les institutions territoriales en profondeur pour se protéger de la volonté populaire. C'est exactement le même mécanisme avec la métropole. La mobilisation dans la durée des « gilets jaunes » est la preuve que les classes populaires,

L'abstention record aux élections régionales et départementales de juin dernier et la faible représentativité des exécutifs locaux doivent provoquer un électrochoc : il faut vraiment décentraliser et simplifier pour faire face aux velléités de toute-puissance de ce que certains ont qualifié de « monstropoles ». C'est pourquoi je voterai cet amendement de repli, qui est en réalité un amendement d'ouverture aux élus locaux, en réattribuant les nombreuses compétences de proximité aux municipalités.

Nombre d'élus communaux dont le seul parti est l'intérêt de leur commune et de ses habitants m'ont fait part de leur consternation devant le dépouillement de leurs compétences en faveur de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, au bénéfice des villes qui y sont majoritairement représentées, notamment Marseille que je qualifierai de tonneau des Danaïdes. Car, si je suis Marseillais, je ne m'enferme dans aucun égoïsme et je tire les enseignements de six années d'agitation métropolitaine stérile qui n'ont servi à rien ou à pas grand-chose, si ce n'est au racket financier de 91 communes au profit d'une seule, Marseille, et au braquage de prérogatives communales au profit d'une structure impotente. Je reste fidèle à mes convictions et je milite pour la suppression de cette métropole, qui aurait pu être une réalité économique, mais qui n'est qu'un mammouth administratif de plus, d'une lourdeur et d'une lenteur handicapantes, éloignant les citoyens de la décision, accentuant la complexification, la dépense publique et le clientélisme, et étouffant les petites communes. Ainsi, la délégation de compétences de la métropole vers les communes prévue par cet article ne peut être limitée au 1 janvier 2024 comme vous le prévoyez. Les délégations de compétences doivent devenir la norme, et non l'exception ; elles doivent être élargies et non contenues. C'est l'esprit de la décentralisation voulue par votre texte. Rien ne justifie donc cette limite dans le temps. De plus, les communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne veulent pas laisser leur compétence voirie à la métropole : il faut qu'elles puissent en conserver la maîtrise. l'ancien préfet des Bouches-du-Rhône, Pierre Dartout, a remis un rapport dont les conclusions préconisent de rendre aux communes leurs compétences de proximité. La métropole d'Aix-Marseille-Provence représente près de 2 millions d'habitants : chacun d'entre eux est confronté quotidiennement à une situation particulière qui revêt une grande importance pour son cadre de vie. Pour assurer l'aménagement et l'entretien de tant de rues, de ruelles et de voies, il faut laisser la compétence voirie à l'échelon le plus subsidiaire. Et cela est valable pour toute compétence de proximité. On se souvient aussi du rapport d'information du Sénat de juin 2019 soulignant le sentiment de dépossession grandissant que ressentent les élus municipaux envers leur intercommunalité. Il y a là une grande part d'explication à l'abstention. Afin de rendre au plus vite leur liberté, et donc leur pleine efficacité, aux communes, je vous propose donc, mes chers collègues, de supprimer de cet article la mention « jusqu'au 1 janvier 2024

Madame la ministre, je salue votre volonté, annoncée dans l'objet de votre amendement, de permettre aux communes de la métropole d'exercer des compétences de proximité « lorsque leur exercice à cet échelon contribue à une grande efficacité de l'action publique

de mettre fin de manière unilatérale aux conventions de délégation conclues avec les conseils de territoire. Le second permet à la métropole de déléguer à ses communes membres l'exercice de compétences qu'elle est censée exercer. La métropole d'Aix-Marseille-Provence est née en 2016 d'un regroupement de six intercommunalités. Cependant, un peu comme à Paris avec les établissements publics territoriaux, le périmètre des anciens EPCI a été conservé pour créer des conseils de territoire qui exercent encore aujourd'hui de larges compétences déléguées par la métropole. Ces délégations sont nécessaires à son bon fonctionnement. Nous proposons donc, par cet amendement, de supprimer l'organisation obligatoire d'un débat sur les délégations de compétences. Les conseils de territoire constituent un niveau de proximité plus satisfaisant que la métropole, et nous ne voyons pas pourquoi ces délégations devraient être remises en cause obligatoirement.

d'un réexamen par le conseil de métropole trois ans après son renouvellement. Par cet amendement, nous proposons que le débat sur la fin desdites délégations de compétences entre la métropole et les territoires se déroule seulement à la demande de l'ensemble des conseils de territoire. Madame

bornes de rechargement des véhicules électriques, voirie de proximité, aires et parcs de stationnement, tourisme, zones d'activités, eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines, mobilier urbain, ainsi que tous les accessoires de l'espace public -sont rendues, avec leur accord, aux communes. Un décret en Conseil d'État définit les caractéristiques opérationnelles, ainsi que le critère de proximité afin d'assurer la cohérence de cette répartition avec l'objectif et les compétences structurantes et stratégiques de la métropole.

reprend les conclusions du rapport Dartout. Il répond aux attentes des maires concernant le retour de compétences de proximité et il ne bloque aucunement la situation.

doivent définir la répartition des compétences entre les différents échelons de la métropole d'Aix-Marseille, à savoir la commune, le conseil de territoire et la métropole en tant que telle.

Madame la ministre,

Nous devons agir sans plus tarder pour permettre à ce territoire d'exercer ses compétences au bon niveau, entre communes, conseils de territoire et métropole. Et j'ai bien entendu l'avis de M. Benarroche sur les conseils de territoire ... Je vous propose donc de continuer à y travailler ensemble dans le cadre de la navette. C'est pourquoi, mais

Sur le fond, j'étais de ceux qui, lors de la première délibération, ont voté contre le transfert à titre expérimental des routes nationales aux régions.

Conformément à l'article 43, alinéa 5, du règlement, lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui présente un nouveau rapport. La commission est-elle prête à présenter son rapport ?

explication de vote. J'entends bien que Mathieu Darnaud, le rapporteur, « tape » sur les socialistes pour essayer de reconstituer la majorité qu'il n'a pas obtenue lors du premier vote ; c'est de bonne guerre.